La séance est reprise. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable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 Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 31. L'amendement n° 177 rectifié,

Cet amendement est contraire à la position de la commission. Les jurys et instances de sélection de la fonction publique doivent être « composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes Depuis le 1 janvier 2015, la proportion minimale de personnes de chaque sexe est fixée à 40 %. Cette proportion est difficile à respecter dans certaines filières, compte tenu d'une trop forte représentation de l'un ou l'autre sexe- je pense aux infirmières.

selon nous, une trop grande rigidité, surtout pour les concours organisés sur plusieurs sessions par an. Par ailleurs, rien n'empêche de procéder à une alternance plus rapide lorsque cela est possible. L'avis est défavorable. Quel est l'avis L'avis est défavorable pour les mêmes raisons. J'ajoute que nous avons un objectif de professionnalisation des jurys, notamment pour intégrer un certain nombre de critères. J'évoquais, avant la suspension, la question de la lutte contre toutes les formes de discrimination et celle de la stabilité, au-delà de la répartition que vous évoquez, madame la sénatrice. Mais votre amendement aurait aussi des conséquences sur la stabilité des jurys et le rythme de renouvellement. Un rythme trop rapide, s'il était imposé, empêcherait la professionnalisation et l'intégration des critères que nous souhaitons

L'article 32 supprime, dans les trois versants de la fonction publique, le jour de carence en cas de congé maladie lié à une grossesse, pour prendre en compte l'état de vulnérabilité de la femme enceinte. Cette disposition est une bonne nouvelle pour les femmes enceintes. Mais nous regrettons que le Gouvernement considère que les autres fonctionnaires ayant des arrêts maladie n'ont pas de motifs de santé légitimes et préfère ainsi stigmatiser les agents publics. Le rapport publié le 13 juin dernier par deux députées du groupe La République En Marche, Cendra Motin et Valérie Petit, sur la réintroduction en 2018 du jour de carence en cas d'arrêt maladie des fonctionnaires n'a pas permis d'établir de corrélation avec la baisse du nombre d'arrêts maladie. d'euros d'économies avec le rétablissement du jour de carence, en 2018, cette mesure a rapporté « seulement » 96 millions d'euros. Je rappelle les résultats de l'enquête de l'Insee de novembre 2017 sur l'impact du jour de carence dans la fonction publique d'État entre le 1 janvier 2012 et le 1 janvier 2014 et le 1 janvier 2014 : sur une semaine donnée, « le jour de carence n'a pas modifié la part d'agents absents pour raison de santé ». La prévalence de ces absences a évolué de la même manière dans le secteur privé et dans la fonction publique d'État. En revanche, ce qui a changé pour les fonctionnaires, c'est la durée de ces arrêts : il y a moins d'absences courtes et davantage d'arrêts longs. Le jour de carence n'a pas eu d'impact sur les absences d'une journée, car au lieu d'aller voir le médecin les agents ont pris une RTT ou un autre type de congé. Avec ce système, comme le délai de carence coûte cher, les agents viennent travailler en étant malades, ce qui peut finir par dégrader

Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement va au-delà de l'équilibre trouvé lors de l'accord du 30 novembre 2018 entre les représentants des employeurs publics et les syndicats de fonctionnaires. L'article 29 prévoit déjà qu'en cas de déséquilibre constaté entre le rapport femmes-hommes des promus et le rapport femmes-hommes des promouvables, les plans d'actions devront préciser les actions mises en oeuvre

une réserve, toutefois, sur son application et sa coordination avec une mesure adoptée dans le cadre de la loi relative à la programmation militaire, la LPM. Peut-être pourrez-vous nous éclairer, monsieur le secrétaire d'État ? Lors de l'examen de la LPM, notre objectif était double : éviter les ruptures de carrière en maintenant l'engagement et en permettant une conservation des droits d'avancement, et poursuivre l'objectif de développement de la réserve. Nuance importante, ce droit à l'avancement se calcule au prorata des jours d'activité au sein de la réserve, soit en moyenne 35 jours par an et par réserviste. Dans quel cadre s'intègre donc la mesure de l'article 33 ? Vient-elle en supplément ou en substitution de ce que nous avions voté dans le cadre de la LPM ? Dans le second cas, la mesure resterait une avancée majeure pour les militaires, mais pourrait poser un problème pour la réserve. En effet, quel serait l'intérêt pour un militaire de poursuivre son engagement au sein de la réserve opérationnelle, si cela conduit à réduire ses droits en matière d'avancement de carrière ? Notre groupe a émis des réticences sur l'utilisation actuelle importante de la réserve, qui est venue compenser les manques d'effectifs. C'est notamment le cas au sein du service de santé santé des armées. Le dévouement de ses personnels est énorme et leur travail, d'excellence, est reconnu par nous tous. Mais la situation reste très tendue, le service est en sous-effectif chronique, malgré l'apport des réservistes. C'est pourquoi il me semble que, si nos craintes étaient confirmées,

dans la limite de cinq ans au cours de la carrière. Le congé pour convenances personnelles, qui correspond à la disponibilité pour les fonctionnaires, ouvre droit à la prise en compte au titre de l'avancement et des services effectifs, toujours dans la limite de cinq ans au cours de la carrière. cours de la carrière. Le congé parental et le congé pour convenances personnelles, en cas de combinaison successive de ces deux dispositifs, sont pris en compte au titre de l'avancement et des services effectifs dans la limite de cinq ans. Par ailleurs, s'agissant du congé pour convenances personnelles pour élever un enfant, dans le cadre du congé similaire de la fonction publique, l'âge de cet enfant sera fixé par décret en Conseil d'État. La rédaction retenue par la commission ne correspond pas à un tel dispositif. En outre, elle supprime les conditions de réintégration du militaire et le quatrième alinéa de l'article L. 4138-16 du code de la défense, qui concerne un congé pour convenances personnelles spécifique aux militaires, car jumelé avec un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. prévoit, à ce titre, les modalités de prise en compte de certaines durées de service dans la réserve opérationnelle. Ce congé pour convenances personnelles assorti d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, spécifiquement créée par la LPM de juillet 2018 pour répondre aux besoins des armées dans le cadre du maintien des compétences rares ou concurrentielles, est un dispositif différent du congé ordinaire pour convenances personnelles pour élever un enfant. En effet, dans cette position de non-activité, le militaire recouvre ses droits à l'avancement au prorata du nombre de jours d'activité accomplis sous contrat d'engagement à servir dans la réserve. Ses conditions d'application ont été déterminées par décret en Conseil d'État.

secrétaire d'État. La commission des lois a voté la création d'un corps de fonctionnaires de l'État pour l'administration de la Polynésie française. Or l'article 1 de la loi du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'État pour l'administration de la Polynésie française, les CEAPF, donne compétence au pouvoir réglementaire pour créer les corps ressortant de ce cadre juridique particulier, y compris ceux relevant de la catégorie A. Il nous semble donc qu'il n'y a pas lieu de maintenir cette disposition législative, puisqu'elle relève du domaine réglementaire. Quel est l'avis de la commission ? de la commission ? Cet amendement du Gouvernement revient sur un apport de la commission des lois concernant les corps de fonctionnaires de l'État pour l'administration de la Polynésie française.

Sauf dans l'éducation nationale, les corps de CEAPF « s'arrêtent » à la catégorie B. Les intéressés doivent donc venir en métropole passer des concours et demander, quelques années plus tard, leur mutation pour revenir en Polynésie. La commission a donc posé ce sujet sur la table et propose de mieux reconnaître le rôle des CEAPF. Nous tenons à cette disposition d'équité par rapport à leurs collègues de métropole. L'avis est défavorable. La parole est

du Sénat cet après-midi pour rejeter cet amendement. Merci pour la Polynésie française est à M. le secrétaire d'État. L'invitation est tentante, et l'argument peut porter ! Je maintiens l'amendement pour une seule raison. Je ne nie pas, madame la sénatrice, qu'il y ait une nécessité ; je dis que cela relève du domaine réglementaire et qu'il faut y travailler. Au risque

à faire prendre en compte l'ancienneté des collaborateurs parlementaires dans les conditions d'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale. Il avait d'ores et déjà été adopté par notre assemblée lors de l'examen du projet de loi pour la confiance dans la vie politique. Comme il n'avait pas prospéré, nous souhaitons qu'il soit repris pour aller à son terme.

de la commission ? Ces deux amendements visent à ouvrir les concours internes des trois versants de la fonction publique aux collaborateurs parlementaires et aux collaborateurs de groupe. Cette disposition n'a pas été retenue par la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour la confiance dans la vie politique. Aujourd'hui, les collaborateurs peuvent se présenter aux concours externes et aux troisièmes concours. Ils sont, en effet, sous contrat de droit privé, et non de droit public. Leur ouvrir, en outre, les concours internes pourrait soulever une difficulté sur le plan constitutionnel : ils seraient les seuls à pouvoir se présenter à trois catégories de concours. La situation serait également déséquilibrée par rapport aux apprentis, aux candidats issus du milieu associatif et même aux élus locaux, qui peuvent seulement se présenter au troisième concours.

Les collaborateurs parlementaires étant assujettis au droit privé, une telle extension ouvrirait l'accès au concours interne à des contractuels de droit privé ; cela aurait pour conséquence

était « difficilement contestable que nos collaborateurs concourent au service public de la législation et du contrôle de l'action du Gouvernement ». Il y a là une forme

Didier Marie, pour explication de vote. qui exercent une mission de service public à nos côtés, pour améliorer le travail législatif, d'avoir la possibilité d'intégrer la fonction publique territoriale. Cet amendement

type d'emploi, en faveur d'une intégration dans la fonction publique territoriale. Cela nous semble raisonnable. À défaut, il faudrait remettre sur le métier la question du statut des collaborateurs parlementaires, une revendication

Il vise à permettre aux agents contractuels de droit local en poste dans les administrations françaises à l'étranger d'accéder à la fonction publique française par le biais des concours internes. Depuis le 1 janvier 2017, ces personnes n'ont plus la possibilité de se présenter aux concours internes d'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C cette situation résulte d'une décision prise lors du précédent quinquennat. L'accès aux corps de fonctionnaires des catégories A, B et C par le biais des concours internes est donc désormais réservé aux agents publics. Cette situation est d'autant plus paradoxale que les concours internes sont ouverts aux personnes qui ont accompli des services au sein des administrations, des organismes et des établissements des autres États membres de l'Union européenne ou des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Le Gouvernement a récemment pris des mesures réglementaires pour autoriser les recrutés locaux à se présenter aux concours dits « de la troisième voie ». Ces mesures vont dans le bon sens, mais nous constatons que le nombre de places offertes à ces concours est inférieur au nombre de places offertes aux concours internes. De plus, la troisième voie est ouverte aux personnes disposant d'une expérience professionnelle dont la durée est plus longue que celle qui est exigée pour pouvoir se présenter au concours interne. Par ailleurs, les textes réglementaires déjà publiés ne concernent que les agents de catégorie C. Pour toutes ces raisons, nous proposons d'ouvrir les concours internes, en sus des troisièmes concours, aux recrutés locaux. Nous souhaitons ainsi permettre aux corps de fonctionnaires du ministère de l'Europe et des affaires étrangères de bénéficier de l'expérience et des compétences acquises par ces agents de droit local, qui jouent actuellement un rôle central dans le fonctionnement des postes diplomatiques et consulaires, des instituts culturels et des établissements scolaires français à l'étranger. Quel est l'avis de

de conforter ces déclarations et ces actions du Gouvernement en faisant figurer dans la loi le principe de l'ouverture des troisièmes concours aux recrutés locaux. Quel est l'avis de la commission ? L'amendement n° 271 rectifié , présenté par Mme Jacky Deromedi, vise à ouvrir les concours internes de la fonction publique aux contractuels recrutés par les services de l'État à l'étranger. On se heurte au même problème que précédemment, puisque, pour beaucoup, ce sont des contrats de droit privé.

pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ma volonté d'ouvrir les concours de troisième voie aux agents recrutés en droit local. Un décret du 21 mai 2019 permet cette ouverture pour la catégorie C, et un décret relatif

Un sentiment de déracinement se fait alors jour, qui nuit à l'exercice de leurs missions d'intérêt général. L'expérimentation que nous proposons ne requiert pas de moyens supplémentaires, dans la mesure où des concours déconcentrés existent déjà. Il s'agit donc de rapprocher la gestion des ressources humaines des agents, et de fluidifier les carrières. Vous conviendrez avec moi que cela s'inscrit tout à fait dans la perspective politique défendue par ce gouvernement dans le cadre de ce En effet, de nombreux agents ultramarins attendent pendant des années leur mutation ; avec une telle expérimentation, ils pourront plus aisément

de la commission ? Cet amendement tend à permettre l'organisation de concours à affectation locale dans la fonction publique d'État. Il s'agit d'un sujet important ; nous l'avons bien perçu lorsque nous avons entendu les représentants syndicaux de la Polynésie française, en compagnie de notre collègue Lana Tetuanui. Toutefois, cet amendement me semble satisfait par l'article 33 du projet de loi, inséré dans le texte à l'Assemblée nationale. En effet, l'alinéa 4 de cet article permet de connaître en amont le territoire dans lequel les candidats seront affectés en cas de réussite aux concours. L'article 33 est même plus large que l'amendement de nos collègues,

d'une affectation locale ; ainsi, les lauréats du concours auront la garantie d'être affectés dans la région pour laquelle ils ont postulé. Cela nous paraît plus protecteur et cela évite de créer une compétence, qui n'existe pas aujourd'hui, au bénéfice des plates-formes régionales des ressources humaines de l'État, qui sont des structures très légères et qui, dans la quasi-totalité des régions, ne seraient pas en capacité d'organiser des concours nationaux à un échelon déconcentré. Ainsi, au bénéfice de l'article 33 , qui, comme l'a dit Mme la rapporteur, couvre l'intégralité des concours de toutes catégories- ce qui n'est pas le cas de l'amendement défendu -, je demande le retrait

Cette expérimentation prévoyait la possibilité de recruter directement jusqu'à 30 % du nombre maximal de postes qui peuvent être pourvus ; cela permettait au ministère des armées de faire face à des difficultés de recrutement, essentiellement liées à des questions d'attractivité des territoires d'affectation dans le cadre de concours nationaux.

Jusqu'au 31 décembre 2022, ces emplois pourront être pourvus, dans six régions pilotes, par une commission de sélection ; il s'agit donc d'une dérogation au principe du concours. La loi de programmation militaire a limité le nombre de personnes recrutées par cette voie à 30 % du total des recrutements. Au regard des résultats satisfaisants de cette expérimentation, l'amendement n° 491 du Gouvernement vise à augmenter ce plafond à 50 % du total des recrutements. Nous n'y sommes pas opposés,

Cet amendement a deux objets. Le premier est de revenir à la rédaction gouvernementale de l'article 33 pour ce qui concerne l'accès au troisième concours. Nous considérons que la formulation adoptée par la commission des lois risque de restreindre

d'un même grade, les candidats ne peuvent pas figurer sur plusieurs listes des admis à participer, quelles que soient les modalités d'accès au concours visées aux 1° à 3° du présent article.

que les dispositions de ces alinéas constituent une barrière à l'accès au concours ; c'est la raison pour laquelle nous en demandons la suppression. Quel est l'avis de

Si le texte de la commission est adopté, les candidats auront l'interdiction de se présenter simultanément à plusieurs concours permettant l'accès à un emploi de même grade, dans des conditions fixées par décret. Je le précise, cette disposition concerne uniquement les concours dont les épreuves sont organisées le même jour.

a étendu la période d'inscription sur liste d'aptitude à quatre ans. Une mission a été confiée à l'inspection générale de l'administration pour dresser un état des lieux de la situation des lauréats. Le rapport de cette mission a mis en évidence un taux de « reçus-collés » inférieur à 10 %. En ce qui concerne la prolongation de la durée de validité de la liste d'aptitude, les auteurs du rapport indiquaient qu'aucune donnée disponible ne permettait d'affirmer que le phénomène des « reçus-collés » serait corrélé à une durée de validité trop faible de la liste d'aptitude. On peut donc en déduire que l'extension de la période d'inscription sur liste d'aptitude depuis 2016 n'a pas endigué le phénomène des « reçus-collés », toujours estimé à 10 % des lauréats.

Cet amendement vise à permettre au lauréat d'un concours ou d'un examen professionnel de la fonction publique inscrit sur liste d'aptitude pour un certain délai de bénéficier d'une suspension de ce délai pendant la durée de son détachement. Pour rappel, les lauréats d'un concours ou d'un examen professionnel de la fonction publique sont inscrits sur une liste d'aptitude en vue d'être recrutés par un employeur public. Cette inscription est valable deux ans et est renouvelable deux fois pour une année. Au terme de ces quatre années d'inscription sur liste d'aptitude, le lauréat n'ayant pas été nommé dans son nouveau cadre d'emplois perd le bénéfice de son concours ou de son examen professionnel. Dans certains cas, la loi a permis de suspendre ce délai, par exemple en cas de congé de maternité ou d'exercice d'un mandat local. En revanche, cette suspension n'est pas accessible aux agents en détachement, au sein ou en dehors de leur administration d'origine. Ceux-ci doivent impérativement, dans le délai maximal de quatre ans, mettre un terme à leurs missions.

de bénéficier d'une suspension de cette inscription le temps de la durée restante de son contrat de projet. Avec cet amendement, la durée de validité de l'inscription sur une liste d'aptitude pourrait être suspendue pour une durée maximale de deux ans. Dans la mesure où le contrat de projet ne pourra donner lieu ni à une titularisation ni à un contrat à durée indéterminée ultérieur et dès lors que la lutte contre la précarité dans la fonction publique doit demeurer un objectif prioritaire du législateur, cette suspension permettra à la personne concernée

Actuellement, une quarantaine d'agents de la fonction publique territoriale y travaillent en permanence pour le compte de leur collectivité. Cet amendement vise à ajouter à la liste des personnes considérées comme fiscalement domiciliées en France les agents de la fonction publique territoriale et hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. Actuellement, les agents des collectivités territoriales en poste à l'étranger ne sont pas soumis aux mêmes dispositions que les agents de l'État, même s'ils relèvent d'un statut de la fonction publique. De ce fait, ils ne sont pas imposés dans les mêmes conditions que les agents publics en service en France. Leurs revenus de source française sont soumis à des taux forfaitaires de 20 % ou 30 % et ils ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global, alors même qu'ils sont assujettis à l'ensemble des prélèvements sociaux- CSG, CRDS. Cet amendement vise à mettre fin à cette situation.

Jusqu'à présent, cette domiciliation n'existe que pour les agents de l'État. Le développement des instances de représentation des régions françaises à Bruxelles conduit les auteurs de l'amendement à vouloir généraliser ces dispositions.

tend à étendre le régime des agents de l'État prévu au 2 de l'article 4 B du code général des impôts- le CGI -aux agents de la fonction publique territoriale qui résident à l'étranger. Le Gouvernement n'y est pas favorable en l'état pour les raisons suivantes. Le régime des agents de l'État constitue une importante dérogation au principe de la domiciliation fiscale. Ce régime, qui est prévu au 2 de l'article 4 B du CGI, s'applique strictement et ne produit ses effets qu'à l'égard des personnels civils et militaires, fonctionnaires statutaires et employés placés sous contrat de travail avec l'État exerçant leur activité à l'étranger en cette qualité. Les agents des collectivités territoriales et des établissements publics en sont donc exclus, comme le précise la doctrine administrative. Pour autant, les agents des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière expatriés demeurent domiciliés fiscalement en France, s'ils répondent aux conditions de droit commun. En application de l'article 4 B du CGI, sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui y ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, celles qui y exercent une activité professionnelle, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire, et celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. En conséquence, durant leur expatriation, les agents des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière conservent leur domicile fiscal en France, s'ils conservent en France leur foyer, c'est-à-dire le centre de leurs intérêts familiaux, ou s'ils ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

Cependant, lorsqu'ils peuvent justifier que le taux moyen d'imposition résultant du barème français appliqué à l'ensemble des revenus mondiaux est inférieur à ce taux minimum, le taux moyen est alors appliqué au revenu net imposable. En pratique, le contribuable établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen lié à la France par une convention fiscale peut bénéficier du dispositif du taux moyen, en annexant à sa déclaration une déclaration sur l'honneur dans l'attente de pouvoir produire les pièces justificatives relatives à ses autres revenus mondiaux.

est en principe soumise au droit commun de la fonction publique territoriale, même s'il peut y être apporté des dérogations par voie réglementaire. S'agissant des statuts d'emplois, notamment du régime des emplois fonctionnels, ils sont fixés, par décret, par analogie avec les règles applicables à la fonction publique de l'État ou à la fonction publique territoriale selon le cas.

principalement à élargir à la fonction publique de la Ville de Paris les dispositions de l'article 7 qui ouvrent la possibilité de recrutement pour les emplois de direction. L'Assemblée nationale a adopté un amendement permettant de garantir l'application des dispositions de l'intégralité du projet

territoriale. Pour prendre le seul exemple de l'éducation nationale, vous savez comme moi que, malheureusement, un grand nombre de postes ne sont plus pourvus

la question des congés bonifiés, ma collègue Annick Girardin, ministre des outre-mer, aura l'occasion, la semaine prochaine, d'ouvrir une concertation avec les parlementaires et les organisations syndicales pour établir un bilan et mettre en oeuvre les engagements du Président de la République en

est une vieille rengaine, je dirais même un chiffon rouge agité pour dénigrer, voire effacer des pans entiers de notre histoire, au cours desquels des luttes sociales ont été victorieuses. Ces luttes ont permis d'obtenir des garanties collectives afin de ne pas laisser l'individu

Cette philosophie est aujourd'hui appliquée à la fonction publique de manière dogmatique et dangereuse, puisque la stabilité de l'emploi public est le corollaire du temps long qui caractérise l'action publique, l'intérêt général, la permanence et la continuité de l'État. Il serait à ce titre intéressant, puisque cette réforme est un copier-coller des ordonnances Travail, de se pencher plus sérieusement sur les conséquences de ces réformes sur la dégradation des conditions sociales et sur la démocratie sociale. Le nouveau monde que vous voulez nous imposer n'est-il pas en réalité un grand retour en arrière ? La réforme que vous nous présentez est bien plus insidieuse que la suppression pure et simple du statut des fonctionnaires. elle ne supprime pas, mais elle introduit le ver dans le fruit. En effet, la possibilité de recourir à des contractuels à la place de fonctionnaires placés sous un statut protecteur ouvre la voie au dépérissement de la fonction publique telle que nous la connaissons. Qui, demain, voudra passer un concours, alors que le même emploi sera potentiellement accessible par copinage ou complaisance politique, rompant ainsi avec la notion d'une fonction publique de carrière Les ruptures conventionnelles et autres détachements d'office ouvrent parallèlement la voie à la suppression annoncée de 120 000 postes de fonctionnaires, à laquelle vous vous disiez pourtant opposé,

Ils sont nombreux, à l'heure actuelle, à s'exprimer au sujet de leurs conditions de travail ; ils essaient de se faire entendre, mais avec ce projet de loi, force est de constater que le Gouvernement et la majorité sénatoriale ne prennent pas en compte leur voix. Cette réforme au forceps, imposée aux agents contre l'avis unanime des syndicats, dégradera durablement les conditions de travail de celles et ceux qui ont choisi de servir l'intérêt général en s'engageant dans le service public. En agissant ainsi, le Gouvernement ne répond ni aux demandes des fonctionnaires ni à celles des usagers qui sont particulièrement attachés au service public et qui demandent plus de proximité et d'égalité d'accès. Or, comme je l'avais souligné lors de la discussion générale, le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas plusieurs amendements du groupe socialiste ont été adoptés. Les collaborateurs du Président de la République seront désormais contrôlés par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, lorsqu'ils partent dans le privé. Le remboursement de la « pantoufle » sera automatique. La pénalité financière sera obligatoire pour les employeurs publics qui ne respectent pas l'obligation de mettre en place un plan d'action pluriannuel en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La mission sur le handicap que j'ai réalisée avec ma collègue Catherine Di Folco a aussi reçu un écho favorable, même si le Gouvernement ne s'est pas attelé à la mise en oeuvre de l'ensemble de nos propositions. Les sénateurs socialistes seront particulièrement vigilants à ce que ces dispositions ne soient pas écartées lors de la commission mixte paritaire. Cependant, le compte n'y est pas ! L'esprit de ce texte reste particulièrement inquiétant.

Surtout, le Gouvernement, appuyé en cela par la majorité sénatoriale, a démultiplié le nombre de postes sur lesquels les fonctionnaires seront mis en concurrence avec des contractuels, aggravant au passage la précarité de ces derniers.

Derrière cet affaiblissement du statut, c'est l'objectif de suppression de 120 000 postes qui se dessine. Les dispositions de ce texte, en revenant sur les principes mêmes qui constituent la fonction publique, la mettent à mal. Nous nous y opposerons donc et ferons entendre notre voix en commission mixte paritaire pour sauvegarder autant que possible notre service public. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote. vote. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous arrivons au terme de ces débats, qui ont duré presque deux semaines,

je voudrais tout d'abord vous dire que le groupe Union Centriste a particulièrement apprécié l'examen de ce texte. Nous avons apporté un certain nombre de contributions et nous voulons

à la fois leur expérience et un regard tout à fait positif. Je voudrais aussi saluer, monsieur le secrétaire d'État, votre implication dans l'examen de ce texte. Vous vous êtes vraiment attaché à répondre avec précision à l'ensemble de nos préoccupations,

aux gestionnaires de la fonction publique- quelle qu'elle soit, hospitalière, territoriale ou d'État -pour recourir à différents modes de de recrutement et de gestion des personnels. C'est indispensable, parce que- le président Delahaye le sait bien -il est impératif que nous puissions, demain, arriver à une meilleure maîtrise des dépenses publiques. Or une meilleure maîtrise des dépenses publiques, lorsque

Bien évidemment, le Sénat a fait entendre sa divergence avec une certaine opportunité, dont nous avons eu l'occasion de discuter, mais je crois que, sur le champ d'habilitation des ordonnances,

seulement pour sécuriser juridiquement le dispositif, mais aussi, sans doute, pour l'ouvrir davantage au dialogue social, est tout à fait envisageable. De la même manière, en matière de déontologie, nos débats ont montré qu'un consensus entre les deux chambres

prévalu pendant ces deux semaines de débat, alors même que l'examen de ce texte a été particulièrement haché, puisqu'il était un peu casé dans les trous de l'ordre du jour, ce qui ne se prête pas à une discussion

de la haute fonction publique. Il me semble donc judicieux de continuer à nous associer à vos travaux. Je pense que le président Delahaye, qui présidait cette commission d'enquête, partagera cette invitation.

nos remerciements à l'ensemble des participants pour la rigueur et l'intérêt de ce débat, qui s'est toujours déroulé de manière respectueuse et constructive. Le Sénat a réalisé un travail approfondi, malgré le caractère très serré du calendrier et l'engagement de la procédure accélérée. Nous avions déjà adopté 154 amendements en commission. En séance, nous en avons adopté plus de 100, qui viennent du Gouvernement, mais également de plusieurs groupes politiques. Beaucoup d'apports du Sénat font l'objet d'un consensus avec le Gouvernement. Nous pouvons les citer : les fonctionnaires momentanément privés d'emploi, les FMPE ; l'amélioration des procédures disciplinaires ; l'introduction dans la fonction publique du congé de proche aidant la préservation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, présidé par Philippe Laurent ; l'extension des concours sur titres ; l'allégement de la formation des policiers municipaux venant de la police ou de la gendarmerie ; la reconnaissance du mérite collectif. Évidemment, certains points de désaccord demeurent concernant le rôle des commissions administratives paritaires, l'intégration des agents handicapés dans la fonction publique et le financement de l'apprentissage dans la fonction publique territoriale. Ces désaccords sont toutefois peu nombreux au regard de l'ampleur du texte. Nous avons déjà trouvé des compromis sur des sujets très compliqués, comme la prime de précarité ou les FMPE.

Sur le fond, je suis en parfait accord avec ce que vient de résumer parfaitement Mme Catherine Di Folco sur les avancées que représente ce texte texte pour la modernisation nécessaire de la fonction publique. Je me félicite de l'accord majoritaire du Sénat sur les propositions du Gouvernement.

extrêmement constructive, et c'est important à souligner, car cela facilite certainement la capacité des uns et des autres à se retrouver sur différentes positions. Je remercie plus particulièrement les membres de la commission des lois, au premier rang desquels son président, M. Philippe Bas, dont j'ai apprécié la présence à nos côtés et l'implication.

certaines dispositions, avec toute la subjectivité que cela implique. C'est aussi utile pour nous comprendre et pour savoir exactement de quoi nous parlons et comment nous envisageons les choses. Il y a des Il y a des convergences entre ce que souhaite le Gouvernement et ce que votre assemblée a voté. C'est la raison pour laquelle j'avais indiqué, lors de la discussion générale, que, sur plus de deux tiers des dispositions adoptées par la commission des lois, quelle qu'en soit l'origine, le Gouvernement portait un regard favorable et ne les remettrait pas en cause par le dépôt d'amendements. J'ai par la suite indiqué à plusieurs reprises que cette approbation, en tout cas ce regard favorable sur les dispositions adoptées par la commission des lois de votre assemblée, demeurerait tout au long de l'examen du texte, c'est-à-dire y compris dans le cadre de la préparation de la commission mixte paritaire. Ce n'est pas un engagement pour la séance ; c'est un engagement pour l'intégralité du débat. Nous avons pu avancer sur un certain nombre de sujets. Je pense notamment à la question de la prime de précarité, où nous avons trouvé, je crois, une disposition équilibrée permettant aux uns et aux autres de se retrouver, tout en garantissant, et c'était le souhait absolu du Gouvernement, le bénéfice de cette prime aux trois versants, notamment à la fonction publique hospitalière. Madame la rapporteur, vous avez cité de très nombreux points de convergence. Je ne les reprendrai pas pour ne pas allonger les débats, mais je partage vos propos. Je dirai simplement, en écho à votre intervention et à celle de Mme Lavarde, que j'ai pris l'engagement d'associer à

de l'apprentissage ou encore du handicap, pour prendre ces trois sujets, mais nous savons qu'il y en a d'autres, autour de la déontologie ou encore des périmètres d'ouverture ou d'élargissement des conditions de recrutement sur contrat. Je forme le voeu, à mon tour, que le dialogue singulier qui va désormais s'ouvrir entre le Sénat et l'Assemblée nationale, d'abord avec les rapporteurs, puis à l'occasion de la réunion de la commission mixte paritaire

assez essentiel que nous puissions trouver les plus grandes convergences possible. Je pense qu'il va modifier profondément les choses et la vie quotidienne des services et des agents. Je ne crois pas et je ne partage pas l'affirmation selon laquelle il y aurait une remise en cause du statut. Au contraire, je pense que c'est une modernisation. À l'issue de nos travaux, nous devons garder en tête un objectif,

Mes chers collègues, aux termes du premier alinéa de l'article 28 de la Constitution, « le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin Je vais lever la dernière séance de la session ordinaire, qui sera close samedi 29 juin à minuit. À partir du lundi 1 juillet, le Parlement sera réuni en session extraordinaire.